conclues entre la France et ses partenaires.

Nous aimerions partager cet optimisme, mais l'enthousiasme des premières heures suscite à présent de nombreux questionnements. C'est au moment où l'accord politique doit se convertir en accord juridique que les crispations resurgissent, confirme Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique Plus la réforme prend de temps, plus les multinationales procèdent à des négociations qui s'apparentent à du chantage. Nous souhaitons par cet amendement concrétiser le projet initial de l'OCDE : « réattribuer une partie des droits d'imposition sur les grandes entreprises multinationales de leur pays d'origine aux marchés dans lesquels elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, qu'elles y aient ou non une présence physique. » Mais notre proposition, beaucoup plus ambitieuse, ne concernerait pas seulement une centaine d'entreprises réalisant plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ni même plus de 10 milliards d'euros pendant dix ans. Nous n'excluons pas, comme le prévoit l'accord, les industries extractives polluantes et les services financiers réglementés. Nous ne taxons pas seulement les surprofits supérieurs à 10 % du chiffre d'affaires, ce qui conduit à exclure Amazon : en 2019, le taux de rentabilité de ce géant n'atteignait que 9 %, et la part des 13 milliards d'euros de ses profits à redistribuer aurait donc été nulle - et ce, avec votre consentement

Le dispositif proposé entend compenser par une incitation fiscale les handicaps physiques des zones non interconnectées (ZNI), où la production d'électricité est beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, en raison notamment de la petite taille des systèmes électriques, qui ne permet pas de rendre le marché local rentable. Je précise par ailleurs que cet amendement ne contrevient pas au principe d'égalité devant l'impôt, le Conseil constitutionnel ayant toujours affirmé que des situations différentes pourraient être traitées de façon différente. Précisément, les collectivités situées de l'énergie (PPE) spécifiques, en raison de leurs particularités. Leur offrir un cadeau fiscal plus incitatif, afin qu'elles puissent dépasser les contraintes qui leur sont propres, est donc complètement justifié.

écologique, il vise à appliquer un crédit d'impôt plus incitatif aux PME et TPE qui, en dépit des contraintes induites par l'insularité, réalisent des investissements productifs ou de services à partir de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées.

Compte tenu de la situation économique actuelle, après la crise de la covid, lever cette limitation afin d'encourager les entreprises à continuer d'investir serait un signal positif envers les acteurs de l'économie corse.

Le non-cumul du CIIC avec la zone de développement prioritaire constitue aujourd'hui l'un des principaux freins au déploiement de ce dispositif adopté en loi de finances pour 2019. Afin de rendre effective et pleinement applicable cette mesure, il conviendrait de la rendre cumulable avec le CIIC, afin que les effets escomptés en termes de création d'entreprise puissent voir le jour.

bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d'imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à taxer plus fortement les services numériques rendus par les multinationales du numérique, souvent appelées Gafam. Ce sujet fait aujourd'hui l'objet d'âpres négociations internationales. Toutefois, l'attitude non coopérative des États-Unis et la concurrence déloyale exercée par ces acteurs économiques nouveaux sur le commerce français, dans ces temps particuliers de confinement et de ralentissement du commerce physique, rend légitime cette taxation, ne serait-ce qu'à titre transitoire.

du 24 juillet 2019. La France n'est pas le seul pays à avoir mis en place une telle taxe sur les grandes entreprises du numérique. Il s'agit au surplus d'une mesure légitime compte tenu des bénéfices retirés par ces entreprises de leurs activités réalisées sur le territoire national. Les auteurs de cet amendement rappellent que la mise en place d'une taxation à l'échelle internationale de ces entreprises reste à l'agenda d'organisations comme l'OCDE ou l'Union européenne. À l'heure où l'Union européenne est justement à la recherche de ressources propres, l'innovation fiscale

Entre-temps, les entreprises assujetties à cette taxe pourront demander la restitution de l'éventuel écart entre le montant de la taxe acquitté et le montant qui aurait résulté de l'application des nouvelles règles.

réduit notre liberté de réception et emporte avec elle les destructions liées au puits sans fond de la société de consommation. Nous proposons donc de de mettre en place une taxe sur les contrats de publicité et marketing engagés par les entreprises, ainsi que sur le chiffre d'affaires des régies publicitaires, à hauteur de 5 %. Moins de 1 % des trois millions d'entreprises de France ont accès au marché publicitaire.

investies, à rebours de l'urgence écologique et climatique. Dans le détail, nous proposons de supprimer le seuil du chiffre d'affaires des personnes assujetties à cette taxe sur la valeur ajoutée et d'en augmenter le pourcentage. Les sommes ainsi collectées permettront d'abonder le budget de l'État et, pourquoi pas, de financer la transition écologique Monsieur le rapporteur

à un déploiement d'écrans publicitaires numériques extrêmement envahissant et qui constitue un gaspillage scandaleux de ressources naturelles. La transformation de nos villes en gigantesques panneaux publicitaires numériques non-stop est un sujet majeur. projet de loi de finances est aussi l'occasion de légiférer enfin sur cette problématique, car une majorité de Français souhaite voir disparaître

Le produit de la fiscalité du commerce physique s'élève à 47 milliards d'euros, alors même que la contribution fiscale des Gafam ne représente que 67 millions d'euros. Par les taxes locales qu'ils paient, les acteurs du commerce français participent à l'aménagement du territoire, ce que ne font pas la plupart des géants du numérique, notamment les. Le dispositif Le dispositif proposé prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu'un point de retrait ou un établissement du fournisseur présent sur le bassin de vie sont assujetties à une taxe forfaitaire, en fonction d'un barème lié au montant de la commande. Par l'exonération prévue en cas de retrait dans un magasin ou un point relais, l'amendement vise à responsabiliser le consommateur en l'incitant à venir retirer son colis dans un point physique, afin d'éviter une livraison parfois superflue. Pour rétablir une équité fiscale et territoriale, il est prévu également d'exonérer les livraisons effectuées par un opérateur disposant d'un lieu physique marchand sur le bassin de vie. Pour favoriser les jeunes entreprises du commerce, il est prévu d'exonérer la livraison faite à partir d'une petite entreprise au sens des entreprises éligibles au fonds de solidarité. Enfin, afin de ne pas défavoriser les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l'amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans les communes de plus de 20 000 habitants.

la taxe que vous proposez ne concerne que les biens commandés en ligne et exclut les biens commandés par correspondance, sans aucune justification. Elle ne concerne pas non plus les biens livrés par La Poste. Or les règles juridiques de l'impôt ne permettent pas de cibler uniquement un type d'acteurs.

rectifié. Le présent amendement, issu d'une proposition de l'Association des maires de France et de France urbaine, vise à modifier le calcul de l'assiette du droit d'enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

dans un souci d'équité fiscale et de limitation des abus, d'asseoir les droits d'enregistrement, à concurrence du nombre de titres cédés, sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenus par ces personnes morales.

Le Gouvernement a les mêmes réserves que M. le rapporteur. Il rappelle qu'un mécanisme similaire a déjà été mis en place de 2012 à 2014, avant d'être supprimé en raison des difficultés de mise en oeuvre signalées par les opérateurs économiques et l'administration. La réintroduction d'un dispositif proche de celui qui avait été créé de 2012 à 2014 aurait les mêmes effets néfastes sur les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Mais je peux assurer les parlementaires que les services de contrôle fiscal font extrêmement attention aux pratiques de pilotage du passif. Ils disposent notamment de la procédure d'abus de droit fiscal, s'ils constatent que l'assiette du droit d'enregistrement a été minorée dans un but exclusivement fiscal. Pour cette raison, l'avis du

parole est à Mme Sylvie Vermeillet. La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d'impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire. Cette mesure a une double vertu, puisqu'elle contribue à la relance économique et encourage la transition énergétique. Pour cette double raison, son arrêt fin 2021, après une année seulement de mise en oeuvre, apparaît insatisfaisant. Les textes d'application du dispositif n'ayant été publiés qu'en juin 2021, n'ont disposé que de six mois pour se l'approprier. C'est une durée bien trop modeste pour permettre sereinement la réflexion, la prise de décision et le lancement de travaux par les porteurs de projets potentiels. Le présent amendement vise donc à prolonger ce dispositif d'un an. Merci,

: d'une part, agir en faveur de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs et de la consommation d'espaces naturels ; d'autre part, privilégier l'implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés tout en soutenant l'économie locale. Tel est le sens de cet amendement.

à l'État alors que les arguments avancés par le Gouvernement pour défendre une telle réforme ont rapidement été contestés. De tels impôts seraient sept fois plus importants en France qu'en Allemagne

est à M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à annuler la baisse massive des impôts dits « de production » engagée par le Gouvernement l'an dernier, dans un contexte de besoin criant de recettes pour l'État. de revenir sur la diminution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises votée en 2020. Le Gouvernement a réduit les impôts de production, mais sans contrepartie pour l'emploi ou l'investissement. tenu du contexte actuel, il est primordial de maintenir les recettes publiques. Une telle baisse des impôts de production a eu pour conséquence principale d'augmenter la dette publique. La mesure a été décidée sans prise en compte de la situation. Notre Notre groupe souhaite redonner à l'État des marges de manoeuvre en matière de recettes publiques.

Nous ne sommes pas moins raisonnables que vous. Nous avons une autre approche, et je crois qu'elle est plus équilibrée.

La multiplication des cyberattaques s'explique en partie par l'accélération de la transformation digitale induite par la crise de la covid-19. En outre, les ETI sont, pour les trois quarts d'entre elles, des entreprises multisites, présentes à l'international, ce qui augmente d'autant leur exposition à la menace cyber.

qui tend à créer un crédit d'impôt temporaire dédié aux dépenses des PME et ETI en matière d'audit, de prévention et de protection face aux risques cyber. Quel est l'avis de

de dispositifs fiscaux pour permettre un développement économique plus équitable. On ne peut pas parler d'« équité sociale » ou d'« équité économique » dans des pays où la vie est deux fois plus chère et où le chômage est deux fois plus important. Il faut donc des outils fiscaux pour tenter de rééquilibrer.

Vous souhaitez une extension des réductions d'impôt pour le financement des bateaux de croisière, en fixant non pas un taux, aujourd'hui à 20 %, mais- cela s'entend -un montant forfaitaire de 500 000 euros par cabine.

Par cet amendement, il est proposé que le crédit d'impôt pour la réhabilitation de logements anciens soit accordé non plus à l'achèvement des travaux,

Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit un abondement de 6 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 3 millions d'euros en crédits de paiement pour améliorer

vise les ménages plus difficiles à intégrer dans le parc social, il renvoie à un décret le soin de fixer les ressources permettant d'accéder à cette défiscalisation.

d'un amendement de suppression. Nous constatons en effet un véritable dévoiement du dispositif de cession de titres ou d'entreprises. Les différents élargissements prévus par cet article contribuent, une fois n'est pas coutume, à favoriser la concentration du capital dans les mains d'une minorité. La parole est

qui leur permet de bénéficier d'un crédit d'impôt, égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette mesure, qui vise à décliner fiscalement le plan Indépendants, doit encourager la formation des dirigeants de PME, afin notamment de leur permettre de mieux appréhender les transformations profondes de l'économie en général et de leur métier en particulier. Cet amendement tend à doubler le nombre d'heures de formation éligibles au crédit d'impôt, en le passant de quarante à quatre-vingts heures annuelles.

sur cet amendement qui a pour objet de répondre à une difficulté de mise en oeuvre d'une disposition de la loi de finances pour 2020 et qui traite du mécanisme d'apport-cession.

La première, quelle est l'articulation de cet alinéa avec les suivants qui maintiennent la mention des délais de cinq ans et de dix ans en vigueur ?

exonère en principe définitivement l'apporteur de toute imposition. Toutefois, pour lutter contre certains montages de donation-cession, ce report d'imposition est transféré sur la tête du donataire, lorsque celui-ci contrôle la société émettrice des titres transmis à l'issue de l'opération. Ce même donataire est à son tour définitivement exonéré, s'il conserve les titres reçus pendant un délai de cinq ans ou de dix ans, selon les cas. Il me paraît utile de souligner que, s'il y a conservation des titres, il y a exonération.

? À l'occasion de l'examen du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2021, le Gouvernement avait expliqué qu'un tel amendement pourrait créer un différentiel de traitement entre les sociétés de capital-risque et les autres sociétés par actions. Il me semble toutefois que les sociétés de capital-risque sont des véhicules spécifiques ; elles ne peuvent pas toutes être assimilées à des sociétés par actions. En

et le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) pour la rendre véritablement efficace dans l'atteinte de son objectif : réduire la spéculation, en particulier sur les produits dérivés et les transactions de très court terme, terme, appelées à haute fréquence, et ainsi les risques d'instabilité. À l'heure actuelle, les transactions de produits dérivés ont atteint le même niveau qu'en 2007 et les activités de ont même dépassé leur record établi juste avant la crise de 2007. La stabilité financière est donc à nouveau fortement menacée par des flux spéculatifs qui ne favorisent aucunement l'investissement productif. Il est urgent d'encadrer les transactions et de remettre le secteur financier à sa place de simple intermédiaire.

aux transactions intervenant avant le transfert de propriété à l'acquéreur- cette disposition a été votée par le Parlement en 2016. Les transactions intervenant avant le transfert de propriété à l'acquéreur sont les transactions intrajournalières, dites, c'est-à-dire c'est-à-dire dénouées au cours d'une seule et même journée. Elles incluent notamment les transactions à haute fréquence, qui consistent à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers. Les transactions à haute fréquence représentent entre 21 % et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la Bourse de Paris. Élargir le champ de la taxe sur les transactions financières à ces transactions est donc plus que jamais d'actualité. L'amendement a deux objectifs d'une part, dégager des recettes fiscales supplémentaires, notamment en vue d'augmenter les financements pour lutter contre à la fois les inégalités et le changement climatique ; d'autre part, combler les limites de l'assiette actuelle de la taxe,

Cet amendement vise à taxer plus fortement les transactions sur les actions et les produits structurés. La taxe sur les transactions financières française, dite « taxe Tobin », a été instaurée par Nicolas Sarkozy en 2012. Elle a trois objectifs : faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques ; exercer une action de régulation sur les marchés financiers ; initier un mouvement d'adhésion des autres États au projet de taxation proposé par la Commission

les dividendes explosent depuis de nombreuses années au détriment des salaires et des investissements des entreprises, ce qui légitime une telle hausse, au demeurant modérée, du taux de cette

M. Emmanuel Capus. Le présent amendement vise à faciliter le recours aux émissions obligataires pour les associations régies par la loi du 1 juillet 1901. La crise a fragilisé la santé financière de ces organisations, lesquelles recherchent désormais des sources de financements alternatifs afin de poursuivre leurs missions d'utilité sociale, en particulier en cette période de crise sanitaire. Les émissions obligataires permettent de renforcer les quasi-fonds propres et donc de sécuriser la solidité financière des organisations en sortie de crise. Le code monétaire et financier permet à ce jour à certaines associations d'émettre des obligations. Cependant, comme pour toute société commerciale, elles se placent sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers dès lors que le nombre de porteurs est supérieur ou égal à 150. Or, d'une part, les associations ne sont pas des sociétés commerciales comme les autres, dans la mesure où elles ont un but non lucratif ; d'autre part, il est plus facile de réunir plusieurs centaines de petits porteurs que quelques dizaines de gros porteurs autour d'un projet à fort impact social. Par conséquent, le doublement du seuil de contrôle de l'Autorité des marchés financiers paraît adapté à la situation de ces structures associatives. Cet amendement prévoit en outre que, jusqu'au 31 décembre 2022, de manière exceptionnelle et dans le contexte de crise, la souscription d'obligations ouvre droit à une réduction d'impôt, dont le taux de défiscalisation serait égal au taux d'IR-PME, dans les limites imparties aux dons aux associations.

Une évolution réglementaire permet d'ailleurs, depuis juin 2020, de rendre éligibles aux contrats d'assurance vie en unités de compte les obligations émises par les associations ou les fondations.

assurant un service d'intérêt économique général (SIEG) du champ des personnes morales à prédominance immobilière. En effet, les foncières solidaires sont des entreprises qui exercent des activités de logement très social et qui mobilisent de l'épargne solidaire. Si plusieurs formes d'épargne solidaire épargne salariale solidaire, épargne bancaire solidaire, épargne de partage -, la forme la mieux adaptée à la mission de lutte contre le mal-logement est l'investissement direct des particuliers au capital de l'entreprise, c'est-à-dire l'actionnariat solidaire sous forme d'actions ou de parts sociales. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement, dont le taux est fixé à l'article 726 du code général des impôts. Actuellement, les foncières solidaires

par l'autorité publique aux organisations dont l'activité est reconnue d'intérêt économique général. Ce mandat, reconnu par l'Union européenne, permet aux organisations de bénéficier

à l'investissement en actions ou en parts sociales. Cependant, contrairement au dispositif IR-PME-ESUS, la plus-value réalisée lors de la revente de titres de foncière SIEG est soumise à une imposition de 30 %. À titre d'exemple, sur un investissement de 1 000 euros au capital d'une foncière SIEG, la réduction d'impôt est de 250 euros, mais lors de la revente, cet avantage est imposé à 30 %, si bien que l'avantage fiscal net est de 175 euros, ce qui dégrade l'intérêt du dispositif. C'est pour cette raison que je demande l'alignement

En effet, ils bénéficieraient d'abord de la réduction d'impôt sur le revenu, puis d'un montant de plus-value minoré lors de l'imposition, ce qui serait pour le moins exorbitant du droit commun. C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet

IR-PME au travers de deux leviers : rendre éligibles au dispositif toutes les sociétés agréées ESUS, quels que soient leurs secteurs d'activité ; permettre aux sociétés agréées ESUS de faire bénéficier à leurs souscripteurs du dispositif fiscal sur l'actionnariat solidaire au-delà de la durée de dix ans.

alors que ces activités sont exclues pour les entreprises de droit commun. Cet amendement permet de pallier cette différence de traitement et de faciliter le développement des entreprises ESUS. Quel est l'avis de

Je veux aussi rappeler que le cumul d'un avantage fiscal à l'entrée et d'un tarif réglementé de rachat de la production à la sortie est apparu excessif et qu'une telle modification ne pourrait de toute façon entrer en vigueur

de solidarité sur la fortune (ISF) décidée par le Gouvernement ne pouvait se justifier que si elle avait pour effet de stimuler fortement l'économie au point de pouvoir générer des gains en termes d'emploi et de pouvoir d'achat. Rapport après rapport,

La suppression de l'ISF répondait avant tout à des motifs idéologiques. Alors qu'approche la fin d'un quinquennat qui a permis de mettre en lumière le caractère fallacieux de la théorie du ruissellement, le patrimoine des plus grandes fortunes françaises a fortement augmenté. de vie (Crédoc), quatre millions de personnes ont basculé dans une situation préoccupante en raison de la crise sanitaire. Aujourd'hui, alors que l'urgence climatique est grande, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose la création d'un ISF climatique sous la forme d'un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

Comme l'indique le dernier rapport d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital de France Stratégie, la suppression de l'ISF n'a pas eu d'effet sur l'investissement. Il se réduit donc à un dispositif destiné à enrichir les contribuables les plus aisés, dont les habitudes de consommation sont par ailleurs les plus polluantes. Face au double constat de l'inefficacité macroéconomique et de l'injustice sociale et environnementale, cet amendement vise à instaurer un ISF climatique. En tant qu'outil de justice climatique, ce nouvel ISF se distingue de l'ancien sur trois plans. D'abord, un nouveau barème d'imposition associé à des taux plus progressifs est introduit pour assurer une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés. Ensuite, un ensemble d'exonérations bénéficiant aux contribuables situés à l'extrême sommet de la distribution des richesses est supprimé, notamment l'exonération sur les biens professionnels, déduction faite d'un abattement de 2 millions d'euros.

conduisent à un taux d'imposition ISF effectif inférieur à 1 % du revenu économique des 0,001 % les plus aisés. Autrement dit, l'extrême sommet de la distribution des revenus échappait largement aux effets de l'ISF et se trouvait, de fait, encouragé à poursuivre un mode de vie particulièrement polluant. Comme le souligne une étude publiée en janvier 2019 dans la revue scientifique, au niveau mondial, le mode de vie des 0,5 % les plus aisés émet autant de CO2 que celui des 50 % les plus pauvres. Dans la même veine, l'économiste Lucas Chancel montre que les 1 % les plus riches émettent 17 % des émissions totales de CO2. L'urgence climatique et sociale exige de mettre fin au dysfonctionnement fiscal en faveur des ménages les plus aisés.

Il vise à réaligner la fiscalité énergétique sur les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues par la stratégie nationale bas-carbone, en intégrant un élément de justice environnementale fort, susceptible de répondre à l'exigence de transition juste édictée en préambule de l'accord de Paris. Une meilleure répartition entre la contribution budgétaire des ménages et leur empreinte carbone permet de contourner les difficultés que pose l'augmentation de la contribution climat énergie (CCE), taxe carbone régressive, en termes de justice sociale, comme l'a montré l'épisode des « gilets jaunes Il s'agit d'organiser un partage de l'effort plus juste au sein de la société. En effet, il apparaît que le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres. À elles seules, les émissions de gaz à effet de serre associées au patrimoine financier détenu par les ménages assujettis à l'ISF en 2017 représentent environ un tiers de l'ensemble des émissions associées au patrimoine financier des ménages français. Cet ISF climatique vise à améliorer l'acceptabilité sociale de la transition énergétique.

Une stratégie indubitablement antiéconomique consistant à vendre un appartement aujourd'hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yacht permet d'échapper à l'IFI. Seraient notamment inclus dans l'assiette de ce nouvel impôt les résidences principales, les immeubles non bâtis, les liquidités et placements financiers assimilés, les biens meubles corporels, les actifs numériques ou les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n'en est ni l'auteur ni l'inventeur. Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l'objectif d'encourager l'investissement productif. Pour rappel, le présent amendement a déjà été adopté par le Sénat sur l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, avec cependant une entrée en vigueur différée au 1 janvier 2021. La présente rédaction prévoit, quant à elle, un remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive dès 2022.

qui ne peuvent pas être considérés comme des moteurs premiers de la prise de risque et des soutiens directs à l'économie. Le présent amendement tend à assimiler aux biens énumérés dans l'actuelle assiette de l'IFI les liquidités et les contrats d'assurance vie investis en unités de compte, c'est-à-dire en actions d'entreprise.

Mme Sophie Taillé-Polian. Plus le patrimoine est mobile, plus les détenteurs de ces actifs sont en mesure d'échapper à l'impôt. Une série d'études réalisées par des économistes montre que les plus aisés utilisent le changement de résidence fiscale dans le but d'éviter l'impôt. Afin de garantir que chaque citoyen s'acquitte de sa juste part d'impôt, cet amendement remplace le domicile fiscal par la nationalité, en tant que critère déterminant de l'assujettissement à l'impôt en France, et supprime les abattements. Ainsi, changer de domicile fiscal équivaudrait à renoncer à la nationalité française. En suivant la législation en vigueur aux États-Unis, ce dispositif réduit la possibilité d'éviter l'impôt par la mobilité résidentielle. De plus, en suivant les travaux des économistes Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, cet amendement introduit une véritable à hauteur de 40 % du patrimoine net de tout contribuable disposant d'un patrimoine net supérieur à 40 millions d'euros qui renonce à sa nationalité.

ce dispositif, un résident français qui transférait son domicile fiscal hors de France était taxé sur les plus-values latentes qu'il pourrait faire s'il vendait son patrimoine dans les années suivant son départ. Je sais que cette taxe ne rapportait pas des centaines de millions d'euros, mais elle était importante symboliquement. Elle avait également son importance en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Par ailleurs, je ne crois pas que nous ayons eu de la part du Gouvernement un bilan de sa suppression ou de sa quasi-suppression en matière d'attractivité.

l'exonération prévue pour le bénéficiaire qui ne présente qu'un simple document de gestion forestière, et maintenir à 75 % l'exonération pour les bénéficiaires respectant des écoconditions ambitieuses relatives à la biodiversité et à la conservation des puits de carbone forestiers. Sur les amendements

réformée par la loi de finances pour 2019. Conformément à la position constante de la commission depuis lors, je suis défavorable à ces propositions, puisque la réforme de 2018 a remplacé un dispositif

un certificat de garantie durable pour bénéficier de l'exonération

la mise en place du PFU favorisait les plus aisés. Ainsi, les 15 % des personnes les plus aisées obtiennent 83 % du gain total de niveau de vie, avec un gain particulièrement concentré sur les 5 % les plus aisés. France Stratégie, dont on a beaucoup cité le rapport voilà quelques instants, nous dit : « On ne détecte là encore aucun impact sur l'investissement et les salaires parmi les entreprises possédées davantage par des personnes physiques suite à l'instauration du PHU.

: « L'instauration du PFU n'a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié du PFU à connaître une évolution de l'investissement significativement différente de celle des autres. » Le PFU a favorisé l'augmentation et la concentration des dividendes. En effet, en 2017, 0,1 de contribuables percevaient la moitié des dividendes, soit 7,6 milliards d'euros. En 2019, 0,1 % des contribuables en perçoivent les deux tiers, soit, compte tenu de la forte hausse des versements, 14,9 milliards d'euros. Ce dispositif entraîne des inégalités fiscales, une baisse de recettes pour l'État, et il n'atteint pas les résultats pour lesquels il a été créé. C'est pourquoi nous souhaitons supprimer le PFU, dans un souci de plus grande justice fiscale et sociale. C'est un amendement identique de suppression du PFU. Cette est injustifiée. Il n'y a aucune raison pour qu'à revenu égal les détenteurs de revenus du patrimoine paient moins d'impôt que les salariés.

revenus du capital en 2013 s'était en fait traduite par une contraction de la base fiscale, et donc une diminution des recettes fiscales perçues au titre des dividendes. Cette démonstration ayant été faite,

M. Thierry Cozic. L'objet du présent amendement est d'augmenter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Cette contribution ne touche que les revenus annuels supérieurs à 250 000 euros, auxquels est appliqué un taux allant de 3 % à 4 %.

Afin de contribuer à financer les effets de la pandémie, l'Argentine, les États-Unis et le Danemark ont mis en place une taxe sur les hauts revenus. Les sommes récoltées serviront à financer des aides sociales, des PME, l'achat de matériel médical, Monsieur le ministre, le Président de la République n'a eu de cesse de dire que nous étions en guerre. Un bref saut dans l'Histoire vous apprendrait qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, le même genre de mesures ont été prises en Italie, en Autriche, en Hongrie et en Tchécoslovaquie. Au lendemain du second conflit mondial, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et la France ont pris la même voie. L'Histoire est un éternel recommencement, disait Thucydide.

Mme Isabelle Briquet. Nous proposons d'instaurer un prélèvement exceptionnel de solidarité sur les encours d'assurance vie. Ces derniers représentaient 1 812 milliards d'euros en mai 2021, même une faible mobilisation de ces réserves permettrait de financer les mesures de soutien à destination des entreprises et des ménages dont nous avons besoin. Nous proposons donc un prélèvement exceptionnel unique très modéré de 0,5 % sur ces encours au titre de la solidarité nationale. Afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d'assurance vie supérieurs ou égaux à 150 000 euros, par référence aux dispositions déjà existantes en matière d'assurance vie.

nous nous retrouvions sur la philosophie d'une telle mesure, mais que la majorité sénatoriale avait une difficulté avec le seuil, j'indique d'emblée que nous acceptons tout sous-amendement qui viserait à rehausser celui-ci, car il est absolument nécessaire aujourd'hui de tout faire pour mettre en place davantage de redistribution dans notre pays. Madame la sénatrice, j'ai l'impression que vous avez une espèce de trouble obsessionnel avec l'assurance.

qui font individuellement un effort pour se prémunir contre des risques d'accident de la vie ou pour améliorer leur retraite. Il faut

n'a mis aucune conditionnalité, notamment sur le versement des dividendes, à toutes les aides versées aux entreprises.

permet de déduire de l'impôt le montant versé sur ce support dans la limite de 10 % du revenu imposable. Lorsque les personnes récupèrent leur épargne pendant leur retraite, les versements de leur assurance sont évidemment imposés au titre de l'impôt sur le revenu. Jusque-là, tout va bien ; c'était bien prévu ainsi. ainsi. Le problème, c'est qu'il y a une faille dans le mécanisme qui permet d'échapper, dans certains cas, au rattrapage fiscal. Si les fonds versés ne sont pas liquidés du vivant du dépositaire, autrement dit s'il y a suffisamment de revenus à la retraite pour ne pas activer le fond PER, les héritiers, grâce à ce vide juridique, peuvent récupérer les fonds sans avoir à compenser la réduction fiscale initiale.

? L'amendement présenté par notre collègue Bernard Delcros part d'un postulat, selon lequel les sommes qui seraient déduites de l'impôt sur le revenu à l'entrée ne seraient jamais imposées en cas de décès de ses titulaires avant la liquidation du fameux plan d'épargne retraite, ce qui me paraît légèrement discutable, puisque la fiscalité applicable dans ce cas dépend de la nature du contrat de PER. Soit il est sous forme de compte titres, et l'épargne transmise sera incluse dans l'actif successoral, donc soumise aux droits de succession ; soit il est sous forme d'assurance vie, cas que vous avez évoqué,

En outre, la solution proposée est celle d'une imposition à l'impôt sur le revenu, ce qui semble moins adapté qu'un assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit, puisqu'il s'agit de sommes transmises en cas de décès.

a pour objet l'aménagement de la niche fiscale, dite « pacte Dutreil », sur les droits de succession d'une entreprise. L'administration fiscale prend ses responsabilités et vient de conclure, voilà quatre mois, un travail sur cette niche fiscale. Elle indique notamment : « Dès lors que l'ensemble des titres soumis à engagement a été transmis, la direction de la société doit être assurée par l'un des héritiers, légataire ou donataire. » En d'autres termes, une telle condition exigerait que les enfants prennent obligatoirement la direction de l'entreprise. Nous proposons de modifier la logique du mécanisme et de mettre en place, non plus une exonération partielle, mais un abattement en valeur. Un tel dispositif permettrait de favoriser la transmission des petites entreprises, tout en fiscalisant les transmissions de patrimoine professionnel de très grande valeur.

Cette possibilité de triple interposition serait néanmoins restreinte aux holdings hébergeant l'actionnariat salarié. En effet, de nombreux cas d'ouverture du capital de PME ou d'ETI familiales à leurs salariés s'accompagnent de la création d'une holding destinée à héberger cet actionnariat salarié.

L'exonération des droits de mutation à titre gratuit s'appliquerait aux parts de la société détenues par le redevable lorsque cette société possède une participation dans une autre société

Cette situation de décalage fiscal du cadre de la transmission entre la France et ses voisins européens perdure depuis le début des années 2000. Elle constitue un désavantage compétitif majeur qui explique que la France soit aujourd'hui le plus mauvais élève de l'Europe en matière de transmission contre 56 % en Allemagne et près de 70 % en Italie. Ce décalage est d'autant plus préjudiciable que la crise économique liée à la pandémie de coronavirus a fragilisé nombre d'entreprises françaises. Par conséquent, dans le contexte critique que connaît actuellement la transmission d'entreprise dans notre pays, le présent amendement vise à instaurer un pacte de très long terme qui permettrait d'aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission

Il conviendra pour ce faire d'inclure dans cette évaluation les dispositifs temporaires que nous avons pu adopter par le passé ; je pense particulièrement à celui que nous avons adopté en 2020 pour les dons de sommes d'argent sous condition de réemploi.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants. Afin de renforcer l'insertion des jeunes et leur capacité à investir, il apparaît aujourd'hui opportun d'encourager la redistribution intergénérationnelle des patrimoines.

poser les choses avec objectivité, parce que j'ai entendu certains de nos collègues appeler notre attention sur les montants dont on parle.

précité de six à dix ans. Enfin, il tend à rétablir l'actualisation annuelle sur le barème de l'impôt sur le revenu du tarif et des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit. travers de cet amendement, fluidifier la circulation du capital par l'assouplissement des conditions pesant sur les donations, d'une part, en portant la limite maximale de capital transmis à 50 000 euros tous les dix ans et, d'autre part, en supprimant la condition d'âge maximal pour le donateur.

L'absence de réévaluation des seuils et des abattements à la base a aggravé la pression fiscale et de façon importante pour les petites successions. Depuis, force est de constater que la situation est d'autant plus prégnante que l'accroissement des inégalités en France est principalement nourri par la croissance des inégalités patrimoniales. La mesure proposée permettrait ainsi de renforcer la progressivité du dispositif, tout en intégrant notamment le renchérissement des prix de l'immobilier, notamment dans les zones métropolitaines denses, mais aussi sur les littoraux français, renchérissement qui a contribué à alourdir la taxation, au titre des droits de mutation à titre gratuit, de personnes aux revenus pourtant modestes.

75 % de la valeur des propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, garantie qui ne permet pas, de fait, une réelle prise en compte

Sans surprise, je suis défavorable à cet amendement qui vise à alourdir la fiscalité de l'assurance vie. Rappelons que les primes versées après 70 ans sont déjà soumises

On constate ainsi une très forte proportion de dossiers surprimés venant alimenter un secteur hautement bénéficiaire : le ratio entre sinistre et prime est L'objet de cet amendement, déposé par notre collègue Catherine Deroche, est de permettre la création de nouveaux contrats d'assurance dits « inclusifs », souscrits en garantie d'un emprunt professionnel ou pour l'acquisition d'une résidence principale.

de malades ou de personnes vivant avec le VIH, qui nous ont expliqué que l'accès à l'assurance emprunteur est toujours aussi compliqué pour un certain nombre de nos concitoyens. Peut-être le dispositif que nous proposons serait-il difficile à mettre en oeuvre, peut-être ne serait-il pas efficient

amendement vise à moduler le mécanisme de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurance de dommages. Il est proposé de faire passer le taux mensuel d'intérêt de 0,40 %, soit 4,80 % par an, à 0,50 % en 2022,

Je demande le retrait de cet amendement, pour deux raisons. D'une part, le dispositif proposé ne me paraît pas opérant. L'article 6 ouvre la possibilité temporaire d'un amortissement fiscal uniquement

Depuis sa création par le général de Gaulle, le dispositif n'a cessé de faire ses preuves. Alors que la crise économique fait peser de lourdes incertitudes sur l'avenir des entreprises et des salariés, la participation apparaît plus essentielle que jamais. C'est pourquoi il convient d'en renforcer l'attractivité, notamment auprès des entreprises. Le présent amendement vise à renforcer ce dispositif en doublant les montants admis pour cette provision. Quel est présent amendement prévoit que le montant de cette provision peut être égal au montant de la réserve spéciale de participation, contre

sa cible, car son objectif est de développer la participation des salariés. Or le mécanisme de déductibilité de la provision pour investissement n'est plus éligible qu'aux

nos sociétés. Il convient que toutes les mesures d'un plan de soutien massif aux entreprises soient totalement compatibles avec ces conversions, en prenant en compte dans leur gouvernance et dans leurs pratiques des critères comme la transition bas-carbone la régénération de la biodiversité et les problématiques environnementales. L'enjeu est d'accompagner les organisations dans la préparation et l'acceptabilité des projets soutenant la transition écologique.

a trois ans, sous l'impulsion de la commission des finances, nous avions, tous groupes confondus, déposé le même amendement afin de mettre fin à ces pratiques, mais l'Assemblée nationale en avait considérablement réduit la portée. Certes, les opérations les plus simples sont empêchées, mais il suffit que, dans le cadre d'opérations techniques

au travail de son rapporteur général de l'époque, Albéric de Montgolfier. Il y a deux éléments nouveaux. D'une part, pour ce qui concerne les montages internes, il s'agit d'élargir le champ des opérations assujetties à la retenue à la source, avec la suppression du critère de durée de l'opération et l'inclusion des instruments financiers qui, s'ils échappent à la qualification juridique de dividendes, en reproduisent les effets. D'autre part, pour ce qui est des montages externes, l'amendement prévoit que l'établissement payeur applique une retenue à la source nulle sur les versements opérés au profit d'un résident d'un État lié à la France par une convention fiscale.

avant les révélations de la presse, et avant même l'instauration du dispositif adopté en loi de finances pour 2019. Cela a donné lieu à des rappels et à des retenues à la source, assortis de pénalités de 80 % et, dans des cas plus rares, de 40 %.

Selon le Gouvernement, avant d'envisager de faire évoluer ce dispositif, il conviendra de l'évaluer, notamment à la lumière des résultats obtenus par nos partenaires. S'il s'avérait que les moyens mis à la disposition de l'administration étaient insuffisants, le champ et les modalités d'application de ce dispositif seraient alors adaptés en conséquence. qui est de la proposition, portée au travers de ces amendements identiques, visant le schéma dit « CumEx », la question est complexe. En effet, les schémas abusifs s'appuient sur des opérations de prêt ou de cession de titres, qui sont des opérations très courantes de couverture de position et font partie de l'activité normale des marchés, en France comme ailleurs. Il convient donc de ne cibler que les situations abusives dans lesquelles le non-résident évite délibérément la retenue à la source sur les dividendes. Cette condition est la seule permettant d'éviter que la retenue à la source que vous proposez ne soit mise en échec par les conventions.

Il pourrait en être de même pour les navires neufs qui sont financés en dehors d'un crédit-bail fiscal, par exemple par un prêt bancaire classique. Cela serait préjudiciable à la mise en oeuvre du dispositif La contrainte fait également perdre à l'armateur qui pourrait bénéficier du dispositif le bénéfice de la déduction exceptionnelle pour les années restantes après le rachat des parts par l'amateur de la société spécifique d'investissement,

le dispositif, de le rendre rétroactif à compter du 1 janvier 2021 et de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2026.

les émissions et la pollution atmosphérique des navires, qui a été voté en 2018, n'est malheureusement toujours pas opérationnel. D'où la nécessité et l'urgence de faire en sorte que cette mesure entre en vigueur. Tel est l'objet de cet article. Deux modifications adoptées à l'Assemblée nationale risquent de remettre en cause cet objectif et, finalement, de faire perdurer la non-effectivité du dispositif. Il convient donc de revenir sur ces modifications, ce qui est l'objet des amendements n I-25 et I-26, que je porte au nom de la commission des I-25 a pour objectif de faciliter l'incitation à l'acquisition de biens permettant une propulsion auxiliaire décarbonée, principalement

de mon point de vue de manière excessive -le dispositif et contient quelques limites d'ordre juridique. Premièrement, ledit amendement vise à étendre le bénéfice du dispositif aux armateurs qui ont opté pour le régime forfaitaire de la taxe au tonnage. Or cette extension serait inopérante puisqu'on ne peut appliquer une déduction fiscale sur un bénéfice fixé de manière forfaitaire. Deuxièmement, cet

pourrait, me semble-t-il, créer des effets d'aubaine préjudiciables à nos finances publiques. Troisièmement, l'amendement prévoit d'aligner le taux de déduction des équipements rendant possible une propulsion auxiliaire décarbonée sur ceux qui permettent une production principale décarbonée. Pour ma part, je suis attaché à ce que l'on conserve une incitation plus forte en faveur de la production principale décarbonée des navires. Enfin, l'amendement propose aussi que la déduction ne soit plus appliquée sur la durée normale d'utilisation du bien, ce qui est la règle pour ce type de déductions, mais sur seulement trois ans. Pour l'ensemble de ces raisons, et parce que les amendements de la commission permettent de rendre le dispositif effectif et de le renforcer,

en optant pour des avions qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent. Il s'agit, à cette fin, d'introduire un mécanisme de suramortissement fiscal dont le taux est fixé à 30 % pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1 janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Cet amendement s'inscrit dans le cadre des propositions de la Commission européenne du 14 juillet dernier, qui visent à favoriser la mutation des flottes d'aviation civile en agissant dans deux directions : l'emploi des biocarburants ; le renouvellement des flottes pour que les avions soient moins consommateurs de carburant, et donc moins émetteurs

; le plafond de cumul avec les transports en commun, qui bride la capacité du forfait à développer une demande pour l'intermodalité ; le fait que les secteurs public et privé ne disposent pas des mêmes avantages. Exclure le montant annuel de la participation de l'employeur à l'abonnement de transports en commun du calcul de l'avantage fiscal fixé à 600 euros tel est l'objet de cet amendement. La loi Climat et résilience nous a certes permis d'avancer en haussant le plafond de 500 à 600 euros, mais ce n'est pas encore suffisant.

Les navires exploités par des entreprises fluviales bénéficient actuellement d'un étalement de la revalorisation de leurs actifs sur une période de cinq ans. Or un étalement sur une période de quinze ans serait plus favorable au secteur : il permettrait de renforcer la solidité financière des entreprises fluviales et, ainsi, de rassurer leurs créanciers et de faciliter la conduite de leurs investissements. En outre, une telle évolution serait rationnelle au regard de la durée de vie des bateaux fluviaux, soit 70 ans d'âge moyen en France. Le transport fluvial a un important rôle à jouer dans la transition écologique de notre pays. Cet amendement vise donc à donner une impulsion à l'activité fluviale et à ses entreprises. Si vous en êtes

de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, afin de favoriser le renouvellement de la flotte au profit de bateaux plus récents ou plus capacitaires, et donc moins polluants. La limitation de cette exonération à 100 000 euros constitue une exception par rapport à d'autres États européens- Allemagne, Pays-Bas, Belgique -, dans lesquels le régime d'exonération ne prévoit pas de plafond. Le présent amendement vise donc à améliorer la compétitivité du transport fluvial face à la concurrence européenne, d'une part, et face à la route, d'autre part, dans une logique de report modal vers la voie d'eau.

s'appliquerait qu'à partir du 150 kilomètre, pour ne pas défavoriser les circuits courts. Les transporteurs seraient ainsi incités à diminuer les distances de transport ou à privilégier des modes de transports alternatifs, ferroviaires

inférieure à 50 kilomètres par exemple, le pouvoir d'établir une zone à circulation restreinte sur le territoire de leur commune ou de leur EPCI afin de lutter contre la pollution atmosphérique et l'insécurité routière générées par le trafic des poids lourds.

Cette taxe doit aujourd'hui être clairement dotée d'un objectif sous-jacent de décarbonation des transports. Son affectation au financement de solutions alternatives au transport routier répond déjà à une telle logique. La taxe d'aménagement du territoire pourrait également adopter une nouvelle logique d'internalisation des externalités négatives du transport autoroutier, et suivre une trajectoire haussière pour mieux en refléter le coût pollution locale, à l'usure des voies annexes desservant les autoroutes, ou à l'incitation au transport routier, source de 28,5 % des émissions de gaz à effet de serre en France en 2017.

Je ne dis pas que c'est bien- et même, je le regrette -, mais c'est ainsi. L'article 32 du cahier des charges des concessions, tel qu'il ressort de la formulation présentée dans l'annexe 5 du protocole de 2015, stipule qu'en cas d'évolution des impôts, taxes ou redevances de nature à dégrader l'équilibre financier de la concession, des mesures de compensation, notamment tarifaires, doivent être arrêtées pour rétablir l'équilibre initial de la concession. Avant 2015, d'ailleurs, les contrats ne prévoyaient ce droit à compensation

que la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) exonérait l'ensemble des véhicules et matériels agricoles quel qu'en soit leur usage, la taxe à l'essieu « nouvelle formule » n'exonère que les « véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes

dont les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kilogrammes qu'une voiture standard. Durant cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %. Pour donner un ordre d'idée, les SUV sont majoritaires dans les classes C à F, qui émettent entre 121 grammes et 250 grammes de CO2 par kilomètre,

Cette révolution du siècle dernier est le symbole des dérèglements de notre temps, comme la surconsommation, l'étalement urbain, l'abandon des centres-villes, la surutilisation de la voiture. Nous proposons l'élargissement de la taxe sur la création de grands parkings de plus de 2 500 mètres carrés, visant à limiter l'artificialisation des sols.

sur le réseau national non concédé et sur les itinéraires alternatifs du réseau géré par les collectivités locales. Cette taxe s'appliquerait dans le cadre des dispositions de la directive « Eurovignette ». Dans ses considérants, cette directive indique que « dans le secteur des transports routiers, les péages, calculés comme des redevances d'utilisation des infrastructures fondées sur la distance, constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durable, puisqu'ils sont directement liés à l'utilisation de l'infrastructure ». Il s'agit d'appliquer le principe du pollueur-payeur.

afin de limiter, à moyen terme du moins, le transport routier sur des longues distances, qui présente un bilan carbone problématique. Une telle mesure permettrait de réduire la demande de transport routier et, par incidence, d'optimiser le transport de marchandises en favorisant d'autres modes de transport.

que le dispositif ne soit pas trop complexe pour les transporteurs, notamment pour éviter des phénomènes de déport du trafic entre certains territoires.

trouver des solutions pour financer les infrastructures.